amendement prévoit, sur le modèle des sociétés de libre partenariat, que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

une sous-catégorie, bénéficie déjà de l'exonération de la TVA, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En outre, l'exonération de contribution sociale de solidarité des sociétés que vous proposez engendrerait une rupture d'égalité au détriment d'autres organismes de financement.

fixé ici à un ratio de 1 à 13 entre la rémunération la plus faible et la plus élevée, la part de salaire dépassant cet écart type serait non déductible de l'impôt sur les sociétés.

émet un avis défavorable, pour plusieurs raisons. D'abord, par principe, les charges de personnels sont déductibles dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives. Ensuite, l'aménagement des règles fiscales ne permettra pas de limiter le montant des plus hautes rémunérations dans les entreprises, vous le savez, car il existe d'autres dispositifs, comme les retraites chapeaux, les parachutes dorés, lesquels relèvent de la liberté contractuelle des entreprises. Ou alors il va falloir mettre en place beaucoup de dispositifs ... Par ailleurs, votre

7 millions de retraités sont obligés de travailler pour survivre.

Ça a baissé ! Le riz coûte moins cher, c'est vrai ... Cet amendement vise à rétablir le troisième taux majoré de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations de plus de 152 000 euros par an, soit 12 666 euros par mois. Ce cadeau fiscal, qui nous a coûté plusieurs millions d'euros,

Est-ce bien responsable ? On frôle parfois l'indécence ... Cette mesure, qui coûterait entre 50 millions d'euros et 100 millions d'euros par an, avait été prise pour renforcer l'attractivité de la place financière de Paris. On a pensé que le Brexit pourrait inciter certains traders de la City percevant de hauts revenus, mais inquiets par les conséquences du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, à immigrer vers l'Europe continentale. Mais sur la place, il y a aussi Dublin, Francfort. L'Allemagne fait aussi ce qu'il faut pour les attirer. Bref, la logique de la compétition nous mène droit dans le mur.

cela. Vous nous avez alors expliqué que vous connaissiez bien les gens parce que vous aviez géré une entreprise. Or gérer une entreprise, ce n'est pas gérer la France. Franchement, le débat que nous avons depuis ce matin

B du code général des impôts est de réaffecter le produit de cession des titres rapportés dans des activités opérationnelles, ce qui inclut notamment des activités immobilières et des activités financières. Il s'agit donc non pas de remédier à des défaillances de marché afin de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, mais bien de financer l'économie productive de manière générale. De ce fait, les actions de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier sont exclues du champ de ce réemploi. Si le présent article 51 adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit un ciblage sur les PME dans le cadre du nouveau remploi indirect des fonds, c'est dans le but de rééquilibrer cette forme de remploi qui, sinon, pourrait paraître plus avantageuse que le remploi direct. Enfin, concernant les sociétés cibles, le remploi direct est autorisé dans des sociétés européennes opérationnelles. Cela étant, si la souscription en numéraire au capital de sociétés peut bénéficier à l'ensemble des sociétés, en revanche l'acquisition sur le marché secondaire d'une fraction du capital d'une société qui exige que la holding en prenne le contrôle est de fait un mode de remploi fléché vers les PME. Par ailleurs, l'ouverture du remploi aux souscriptions de parts de fonds et de sociétés du capital d'investissement est strictement encadrée. En exigeant de ces structures le respect d'un quota d'investissement de 75 % au titre de sociétés européennes, il s'agit bien de s'assurer que les sommes remployées bénéficient effectivement, et de manière très prépondérante, à des sociétés opérationnelles. Pour toutes ces raisons- nous avons bien encadré le dispositif

-ne nous semble pas conforme au règlement général d'exemption par catégories, et donc à la réglementation européenne. Afin de remédier à ces deux inconvénients, le présent amendement inclut les titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, permet les rachats d'actions dans certaines conditions et, enfin, permet aux fonds

convertibles en actions- OCA -dans le quota de 75 % qui ne correspond pas à l'objectif du dispositif, dès lors que ces actifs obligatoires ne conduisent pas nécessairement, du moins à bref délai, à une entrée au capital des entreprises opérationnelles.

de Philippe Dominati. Compte tenu des différentes transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l'effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l'apport initial, et de la difficulté qu'est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l'obligation d'établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux qui sont initialement apportés. La parole est à

donner un bonus fiscal aux mauvais choix d'investissement. On peut se tromper ; de là à être exempté d'impôts, cela ne me paraît pas forcément une très bonne idée. Aussi, l'avis est défavorable sur ces deux amendements.

La suppression de cette niche fiscale pose un problème, car elle ne traite pas le cas des sociétés en question qui ont été créées voilà plus de dix ans, qui sont en gestion extinctive mais qui n'ont pas encore distribué tous leurs dividendes et ont

: La parole est à M. Serge Babary. Il s'agit, par cet amendement, de favoriser l'investissement dans le capital des PME. La suppression de l'ISF s'est traduite par la suppression de l'ISF-PME, qui constituait un canal du financement de l'amorçage des start-up particulièrement efficace.

de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d''une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME, et ce jusqu'en 2022.

Malgré l'assouplissement de ses conditions d'application, ce dispositif n'avait pas atteint son objectif : son coût annuel s'est chiffré, entre 2008 et 2011, à 2 millions d'euros, pour un nombre de bénéficiaires oscillant entre 2 500 et 3 000. Cela s'expliquait notamment par l'existence d'autres régimes permettant d'atteindre plus efficacement le même objectif. Les dispositifs en faveur des PME, plus incitatifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2012, rendent, de notre

Par ailleurs, le dispositif PEA-PME, mis en place à compter de 2014, vise également à réorienter l'épargne des ménages vers les investissements dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Plusieurs mesures visant à dynamiser ce produit d'épargne ont été adoptées ces dernières années. À cet égard, votre assemblée a adopté, dans le cadre de l'examen du projet

Certes, pendant des années, nous avons eu le sentiment que, par rapport à l'Hexagone, la Corse subissait un préjudice, et les outre-mer, c'était encore autre chose. Par compréhension, et par expérience, et indépendamment de ce que décidera mon groupe, je soutiendrai cet amendement.

d'État. Dès lors que les conventions signées par le ministre de la culture avec les parties emporteront octroi d'une exonération d'impôt, totale ou partielle, il est essentiel que l'administration fiscale ait un droit de regard sur ces opérations qui vont au-delà d'un avis simple. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les conventions soient conclues après avis conforme du ministre chargé du budget. Il s'agit d'un amendement technique.

Cet amendement revient, après avoir été retiré lors de la première partie. Il a été corrigé conformément à ce que souhaitait le rapporteur général. Il s'agit de supprimer une aberration.

qui n'a aucun fondement. Puisqu'il n'y a plus de conservateur des hypothèques, il n'y a aucune raison d'avoir un salaire du conservateur des hypothèques. C'est aussi simple que ça ! Quel est l'avis de

puisqu'il s'agit de mettre un terme à l'exonération de droits lors d'une succession pour le conjoint survivant, dès lors que les époux étaient mariés sous un régime communautaire. Comme l'indique le rapport, la mesure de l'article 1133 du code général des impôts a sans doute perdu une bonne partie de sa pertinence avec la loi TEPA de 2007. Cette loi pour le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat c'était, entre autres travaux, employée à assurer le patrimoine de quelques riches familles en posant un certain nombre de principes une exonération de fait du conjoint survivant et un très large allégement fiscal pour les descendants en ligne directe, grâce à un très sensible relèvement de l'exonération par part. part. Outre les successions, cas évidemment le plus directement évoqué, le dispositif trouvait sa pleine application en cas de donation, offrant ainsi un remarquable outil d'optimisation fiscale à double détente : une fois pour les droits de mutation, et une seconde fois pour l'ISF. De fait, notre pauvre article 1133 perdit une bonne partie de sa substance, le statut de conjoint survivant suffisant pour alléger la contrainte fiscale. On nous dit aussi que la contrainte fiscale qui serait occasionnée est faible, voire peu pertinente. Il s'agit de 32 millions d'euros pour un nombre indéterminé de cas. Donc, nous nous sommes posé la question : pourquoi ? Pour trouver une petite recette de poche permettant de combler un petit morceau du déficit public, madame la ministre, ou pour inciter les personnes concernées à « placer leur patrimoine sous d'autres formes pour échapper à l'imposition future » ? La question induit la réponse. Nous retenons cette dernière hypothèse eu égard à la qualité de la première signataire de l'amendement adopté à l'Assemblée, Mme de Montchalain, qui a derrière elle une expérience de l'assurance vie, du placement dont on ne peut que rappeler tout l'intérêt qu'il recouvre en termes de fiscalité. Mais cela suffit pour que nous puissions vous proposer la suppression de cet article d'opportunité.

de manière générale, à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Ainsi, après de longues années de controverse parlementaire sur la possibilité laissée aux emprunteurs de résilier des contrats d'assurance parfois placés en vente forcée par des établissements de crédit prêteurs, une controverse d'autant plus évidente que la marge commerciale est particulièrement élevée sur ce type de contrat, nous voilà avec une poussée de fièvre.

Or voilà que l'on nous propose de prélever 540 millions d'euros- le rapport, vous me direz si je me trompe, parle de 577 millions d'euros -dans la poche des emprunteurs pour un motif qui nous échappe totalement.

Les emprunteurs deviendraient donc les victimes de la baisse des taux nominaux comme des taux réels, une baisse qui s'explique, notamment- faut-il le rappeler ? -par la faible progression des rémunérations.

Voulez-vous que les ménages soient endettés- il va falloir répondre à cette question ! -, alors que les taux sont bas et que l'essentiel du taux effectif global procède de l'assurance emprunteur majorée de la taxe spéciale

dans sept ans quand tous les contrats auront été renouvelés ; il ne s'agit pas de 500 millions d'euros la première année. En outre, les recettes en résultat seront affectées à compter des impositions établies au titre de l'année 2019 à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil

pour faire plonger un secteur aussi important pour les particuliers et pour les Français, mais aussi pour l'emploi et nos entreprises ? On nous dit que 120 000 emplois vont disparaître l'année prochaine dans le secteur. C'est cela le résultat de la politique que vous comptez mener ? Effectivement,

nous serons unanimes, je le crois, pour soutenir les amendements que nous avons déposés. Il est vraiment grand temps d'entendre que l'accumulation des augmentations de taxes ou de taxes nouvelles n'est aujourd'hui plus acceptable. La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.

Vous ne pouvez pas dire que, lorsque vous taxez une entreprise, quand bien même il s'agit d'une société d'assurance- il est facile d'effrayer le bon peuple avec les sociétés d'assurance ! -, ce n'est pas le consommateur final qui paiera ! Pas vous, madame la secrétaire d'État, pas avec les études que vous avez suivies, pas avec les cours d'économie que vous avez suivis

de particuliers, voire de collectivités, ont souscrit des assurances dommages dans le domaine de la construction auprès de sociétés basées soit au Danemark soit à Gibraltar. Que s'est-il passé ? Ces sociétés ont déposé le bilan,

de 12 % à 25 % le plafond légal de la contribution des assureurs au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, notamment en matière d'accidents de la circulation. Cela procède un peu du même raisonnement que pour les amendements précédents, mes chers collègues. Cet article, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va augmenter de 12 % à 25 % la contribution des assureurs à ce fonds, qui garantit contre les accidents les personnes qui ne sont pas couvertes par une assurance.

indirectement les cotisations d'assurance automobile ne paraît pas être une bonne chose. C'est pourquoi je vous demande de supprimer cet article.

Et les assureurs ne se privent pas de vous le dire, d'ailleurs. Effectivement ! Simplement parce que vous habitez dans le département de la Seine-Saint-Denis : on considère qu'il y a plus de risques que la voiture soit brûlée, volée, qu'un type sans permis vous rentre dedans.

Je veux remercier

Afin de ne pas pénaliser les plus petits exploitants agricoles, nous souhaitons atténuer la dégressivité de l'abattement « jeunes agriculteurs » prévue à l'article 53 du projet de loi de finances. Il est ainsi proposé de maintenir l'intégralité de l'abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n'excède pas le montant net de trois SMIC, soit 43 914 euros, et de 100 % pour l'exercice d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, alors que, dans le projet du Gouvernement, La limite supérieure de bénéfice donnant droit à un abattement n'est pas modifiée : au-delà, et dans la limite de 58 552 euros, soit quatre fois le SMIC, le taux de l'abattement est ramené à 30 % et à 60 % pour l'exercice d'octroi de la dotation. Pour la fraction du résultat qui excède cette limite, l'abattement ne s'applique plus. En outre, il est proposé de renforcer l'attractivité du dispositif pour les petits exploitants qui ont besoin d'un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité. Les jeunes agriculteurs dont le bénéfice est inférieur ou égal à trois SMIC obtiendront, pendant les cinq premières années d'exploitation, un abattement de 75 % de leur bénéfice. Enfin, comme mon collègue, nous précisons que, pour l'exercice d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, le montant total des abattements de 100 % et de 60 % ne peut être inférieur au montant de cette dotation. La parole

du code général des impôts : il s'agit de préciser que les bâtiments destinés à serrer les récoltes, ainsi que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles, sont éligibles à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En d'autres termes, il convient de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.

à une activité de nature commerciale, y compris lorsqu'il est réalisé par un collectif d'exploitants réunis au sein d'une société dédiée, ce qui est fréquemment le cas. Pourtant, la nature juridique du compostage est bien agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situe assurément dans le prolongement de l'activité agricole de chaque associé agriculteur. Comme pour la méthanisation auparavant, et alors même qu'il s'agit d'une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si les matières entrantes sont majoritairement issues d'exploitations agricoles. L'activité de compostage suppose l'exploitation d'un d'un nombre important d'immeubles et d'aménagements fonciers- fosses et silos de stockage, fosses de compostage -aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties.

de leurs effluents d'élevage et, à titre accessoire, trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires. Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, laquelle suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l'activité de compostage agricole, y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l'issue du processus, qui ont une nature qui ont une nature et une destination majoritairement agricoles, soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE, à l'instar de l'activité de méthanisation agricole.

cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles. D'autre part, cet amendement vise à exonérer de la cotisation foncière des entreprises les exploitants agricoles ou sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles pour leur activité de compostage, dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d'exploitations agricoles. Par ses deux volets, cet amendement vise à sécuriser d'un point de vue fiscal les exploitants agricoles qui exercent des activités de compostage et, de fait, à encourager cette pratique : elle permet non seulement une gestion locale des déchets, en limitant les transports, mais aussi une amélioration de la structure et de la fertilité des sols, à travers l'utilisation du compost. Quel

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016. En outre, depuis le projet de loi de finances pour 2017, l'âge minimal ouvrant droit à cette demi-part

au premier chef par la baisse du pouvoir d'achat. Désormais, la grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés

chers collègues, le développement économique des outre-mer nécessite de nombreux outils d'incitation, dont l'aide fiscale à l'investissement, qui est devenue l'un des dispositifs les plus efficaces. La loi de finances pour 2014 l'a profondément modifiée par deux mécanismes nouveaux de crédit d'impôt. Toutefois, leur mise en oeuvre pose problème, car ils sont difficiles à évaluer. En effet, les aides fiscales à l'investissement productif et les aides dans le secteur du logement s'établissent à des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils ont été. Dans un récent rapport, le député Olivier Serva remarque notamment que le montant cumulé de ces aides a baissé de 36 % depuis 2010, ce qui représente une diminution de 445 millions d'euros. L'intérêt du nouveau mécanisme de crédit d'impôt réside essentiellement dans le fait que le versement de l'avantage fiscal est assuré à l'exploitant, sans coût intermédiaire résultant de l'intervention d'investisseurs et de monteurs en défiscalisation. Mais, en conséquence, l'aide attendue par les entreprises est perçue de manière décalée, et ces dernières doivent trouver une solution pour obtenir un préfinancement dans l'attente de cette perception. Sans réponse adaptée quant au préfinancement à taux zéro des investissements, on peut s'inquiéter des effets répulsifs, à terme, du crédit d'impôt,

ce qui les empêche bien souvent d'avoir accès au crédit dans des conditions satisfaisantes. En tout, 65 % des entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. à 2 millions d'euros. Le Livre bleu outre-mer conclut à une demande forte de simplification des dispositions de défiscalisation et de souplesse quant à l'appréciation des conditions de délivrance d'agréments, ainsi qu'à une réduction des délais d'instruction des dossiers.

est, monsieur le rapporteur

est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 W

économique des outre-mer, seuls les restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Le secteur de la restauration étant un vivier d'emplois et un levier touristique important, il est nécessaire d'élargir le bénéfice de l'aide à des restaurants

et la société en commandite simple, ou SCS, et, pour cette dernière, uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires. Ainsi, alors que l'article 199 B renvoie à l'article 217,

Cela leur confère en effet une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié, puisqu'ils sont, dans les faits, des associés passifs ne participant pas à l'activité. L'objectif de cet amendement est d'étendre l'utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d'agrément préalable. La parole est à M. Maurice Antiste, L'objet de cet amendement est d'étendre l'utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d'agrément préalable, le statut d'associé limitant l'engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux au compte courant de la société.

l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ? La différence de statut juridique et fiscal entre les associés commanditaires de SCS et les autres associés de sociétés de personnes justifient leur exclusion du bénéfice de l'avantage fiscal.

Le passage du dispositif de défiscalisation ouvert par les investissements productifs neufs en outre-mer à un dispositif de crédit d'impôt était conditionné à la mise en place d'un mécanisme de préfinancement à taux zéro afin de préserver la trésorerie des entreprises. L'article 55 revient sur cette obligation de préfinancement,

à maintenir l'obligation de préfinancement à taux zéro.

L'Assemblée nationale a limité la restriction imposée par l'article 55 dans sa version initiale en autorisant les schémas locatifs dans lesquels serait présente la Caisse des dépôts et consignations.

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle le crédit d'impôt pour investissement productif est réservé aux investisseurs des

dont l'activité principale relevait de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt. Cet amendement vise à maintenir une cohérence entre les dispositions du projet de loi de finances pour 2019 et celles qui ont été votées dans la loi EROM, en réservant le dispositif du crédit d'impôt aux entreprises qui exercent leurs activités dans un territoire ultramarin, sans restriction sectorielle ou géographique au sein de l'ensemble de l'outre-mer.

aura été multipliée par 3,7 en Guadeloupe ou 3,5 en Martinique. Ces progressions plus fortes qu'en métropole posent de façon aiguë la question de la prise en charge de nos seniors. En Polynésie française, entre 1988 et 2027, le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5,6. Or toutes ces collectivités ultramarines se trouvent déjà en sous-équipement chronique

L'aide fiscale à l'investissement outre-mer s'applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, sous condition d'agrément préalable du ministre du budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés. Il apparaît dès lors possible, et souhaitable, et j'espère que je serai suivi, qu'elle puisse s'appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées, dépendantes ou non, afin de combler un besoin essentiel des populations ultramarines. Quel est l'avis de

aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. En effet, cette exigence introduite, par la voie d'un amendement non débattu, à l'article 21 de la loi la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer se révèle sans aucun lien avec les objectifs visés par le législateur en instaurant des régimes fiscaux d'aide en faveur des départements et collectivités d'outre-mer, ni avec les légitimes exigences en matière d'obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts, droits et contributions qu'il est en droit de requérir des entreprises ultramarines en contrepartie des aides accordées.

en pratique, ce délai n'est que très rarement respecté par les entreprises, en raison de circonstances particulières liées au travail des comptables et des experts-comptables, voire des commissaires aux comptes, ainsi que des retards ou indisponibilités des greffes des tribunaux ultramarins.

du code général des impôts pour circonscrire l'obligation de dépôt aux comptes annuels du dernier exercice social clos. Ainsi, les investisseurs pourront aisément vérifier que l'obligation de dépôt au greffe du tribunal a été satisfaite.

la société effectuant l'investissement et l'exploitant doivent avoir satisfait à l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels un mois après l'approbation d'une part, l'investisseur n'est pas toujours en mesure de vérifier que l'exploitant a bien satisfait à ces obligations et, d'autre part, notamment du fait du fonctionnement des greffes des tribunaux, il peut arriver que l'obligation soit satisfaite dans un délai supérieur à un mois. peut donc se produire entre le fait générateur de la réduction d'impôt, soit la réalisation de l'investissement, et la date à laquelle l'obligation administrative est respectée, parfois pour des raisons extérieures à l'exploitant, à l'investisseur.

à la date du dernier exercice social clos avant la mise en service de l'investissement.

c'est bien à la date de la réalisation de l'investissement, qui est le fait générateur de l'avantage fiscal, que l'entreprise en charge de financement et l'entreprise exploitante qui en bénéficie doivent être à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales.

Il concernerait les logements sociaux de moins de vingt ans, qui, en l'état actuel du droit, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux. en effet, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 C est accordé au titre des acquisitions et constructions d'immeubles et des acquisitions d'immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l'exclusion des réhabilitations d'immeubles. Le parc locatif des outre-mer subit régulièrement les conséquences d'événements climatiques d'ampleur exceptionnelle engendrant d'importants dégâts, comme celui qui a frappé Saint-Martin l'an dernier, sans que l'aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là. Cette mesure serait cohérente

Je comprends très bien le propos de notre collègue : les événements climatiques dramatiques qui ont atteint, en particulier, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Maurice Antiste. Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art dans nos territoires,

Au-delà de leur caractère de propriété privée, les oeuvres d'art sont des trésors nationaux, faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Dans la mesure où l'intérêt public transcende le particulier, le déplacement d'un objet d'art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en oeuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens. C'est pourquoi cet amendement a pour objet d'alléger la fiscalité applicable aux livraisons d'oeuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d'outre-mer. Quel est l'avis de

un certain nombre de dispositifs, y compris de nature fiscale, de soutien à la création ; je pense en particulier à l'achat d'oeuvres d'art par des entreprises et à l'acquisition d'oeuvres d'art destinées aux collections publiques, deux dispositifs fiscaux applicables

Ce crédit d'impôt permettra également aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du parc privé, après passation d'un bail de réhabilitation, de mieux pouvoir engager

dispositif de réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation menés par les particuliers sur leur résidence principale achevée depuis plus de vingt ans. Je ne vois pas très bien ce que

? Il est également défavorable. La réhabilitation du parc privé ancien ultramarin est encouragée, que ce soit par l'avantage fiscal spécifique que constitue la déduction d'impôt outre-mer ou par le régime général de déduction des charges foncières, qui prévoit déjà la prise en compte de certaines dépenses d'impôt.

définition répondrait à un principe simple : les bénéfices réalisés par des multinationales en France doivent être imposés en France. Il n'est en effet pas normal que ces multinationales profitent des infrastructures situées en France pour réaliser des bénéfices, sans contribuer au financement de ces mêmes infrastructures. Par ailleurs, cet amendement a pour objet de prévoir une période transitoire de dix ans,

avis défavorable, pour les mêmes raisons. Madame la ministre,

Cet amendement tend à compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d'impôt sur les sociétés aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d'HLM à l'occasion de ventes de locaux commerciaux, à la condition qu'ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les quatre ans, dans la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

l'avis du Gouvernement ? Le secteur du logement social dispose déjà du dispositif d'incitation, puisque les cessions d'immeubles ayant pour objet la transformation en logements, notamment sociaux, d'immeubles commerciaux ouvrent droit à un taux réduit d'impôt sur les sociétés.

soit nous laissons ce patrimoine s'abîmer et, de toute façon, disparaître ; soit nous laissons faire et, en termes de souveraineté numérique, il se peut que les géants du s'en emparent, ce qui signifie

Cet amendement vise à solutionner les cas de double imposition auxquels sont confrontés certains contribuables à la suite de redressements fiscaux, situation de double imposition que ces contribuables ne comprennent pas. Pour vous donner un exemple, l'administration fiscale qualifie de plus en plus fréquemment une société étrangère qui a réalisé un certain nombre d'opérations en France d'établissement stable, la redresse et l'oblige à s'acquitter de l'imposition en France, à savoir l'impôt sur les sociétés, mais également la taxe sur le chiffre d'affaires qui est réalisé dans notre pays. Or, dans cette situation, la TVA a déjà été acquittée par le client de l'établissement stable en question, ce dernier l'ayant bien entendu obligatoirement autodéclarée. Nous sommes donc bien dans une situation de double imposition, une fois au titre de la TVA sur le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement stable, et une fois au titre de la TVA payée par le client de l'établissement stable. D'après les dispositions actuellement en vigueur, l'administration fiscale n'a pas d'autre choix que de réclamer cette double imposition et ne peut accorder ultérieurement aucune remise gracieuse. En conséquence, cet amendement prévoit d'étendre les pouvoirs de l'administration fiscale en lui permettant, si elle le souhaite, d'accorder des remises gracieuses, dès lors que l'on se trouve dans un cas de double imposition avéré et que, de ce fait, le Trésor ne subit aucun aucun manque à gagner. Une telle mesure augmentera bien entendu la marge de manoeuvre de l'administration dans sa gestion des contrôles fiscaux, ce qui sera de nature à en faciliter le règlement rapide et négocié, évitant ainsi de nombreux contentieux. Aussi, cela améliorera la rapidité des contrôles en permettant l'encaissement immédiat des autres impositions non concernées par les remises. Quel est l'avis

du droit d'asile, qui prévoit que « les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts ». Les dispositions

a retiré la possibilité pour les inventeurs- je parle des personnes physiques -d'imputer sur leurs revenus le déficit constaté lors des frais de prise ou de maintenance d'un brevet excédant les gains tirés dudit brevet. On dit souvent que la France ne dépose pas assez de brevets. Pourtant, certaines personnes physiques en déposent, et je ne vois pas pourquoi on leur supprimerait un avantage

les termes mêmes du rapport, « le dispositif d'exonération proposé est similaire à celui prévu par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2018 pour les " bassins urbains à dynamiser ", dispositif qui concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. « Il est particulièrement regrettable que le zonage régional proposé par le présent article inséré par l'Assemblée nationale intervienne par la voie d'un amendement du Gouvernement, et non par un article initial du projet de loi de finances, qui aurait permis au rapporteur général de disposer d'une évaluation du dispositif et d'un chiffrage précis de ses effets.

en raison notamment de son relief, la Corse connaît une densité de population trois fois plus faible que la moyenne française » ; « son PIB par habitant est inférieur de 5 % à la moyenne de la France métropolitaine, ce qui en fait le troisième plus faible des régions, après les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté au surplus, l'écart du ratio de PIB par habitant par rapport à la moyenne de la France métropolitaine s'expliquerait par la plus faible part de la population occupant un emploi. Le taux d'activité au sein de la population âgée de 25 à 54 ans est inférieur de 6 points en Corse, par rapport à la moyenne de France métropolitaine. » « Ce dispositif d'exonération fiscale vise à remédier au manque de capacités productives en Corse en tendant à inciter les entreprises à s'installer sur l'île. « D'après l'exposé des motifs de l'amendement le dispositif d'exonération fiscale prévu par le présent article vise à accroître " l'attractivité des territoires ruraux et montagneux afin de renforcer leur vitalité socioéconomique " . » Il eût peut-être mieux

de solliciter l'administration pour valider l'éligibilité d'une entreprise ou d'un investissement si le programme ne dépasse pas ce seuil. L'amendement vise simplement à permettre cette saisine par voie de rescrit fiscal.

l'éligibilité d'une entreprise ou d'un investissement si le programme ne dépasse pas ce montant. Le présent amendement vise à rendre possible, pour les entreprises qui le souhaitent, la sollicitation d'une position de l'administration fiscale par voie de rescrit, afin de définir l'éligibilité de leur programme d'investissement. Il s'agit, ainsi, de protéger les investisseurs.

imposés par l'éducation nationale, à travers les choix des conseils d'administration des établissements scolaires. Ainsi, c'est un juste droit d'accès équitable à la culture éducative pour tous les Français que l'on fait vivre.

vise à ouvrir l'éligibilité à la défiscalisation nationale des bateaux de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. C'est une grande avancée pour les collectivités d'outre-mer, mais les conditions édictées sont trop restrictives pour permettre le développement réel du secteur de la croisière en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Je défendrai donc quatre amendements, que nous portons avec mes collègues polynésiens, Mme Lana

Il prévoit des conditions d'exploitation des navires quasi exclusivement sur la zone économique exclusive, ou ZEE, en gardant un pourcentage minime de sortie hors de cette zone, notamment pour tenir compte des spécificités géographiques de la Polynésie française.

? Il nous semble que le secteur de la navigation de croisière, qui est en plein essor, va bénéficier pour la première fois d'aides fiscales du gouvernement polynésien, en plus de la défiscalisation nationale qui s'appliquera dès 2019. La mesure adoptée à l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, représente déjà un geste fort de soutien en faveur de la navigation de croisière dans les outre-mer. Il nous paraît difficile d'assouplir davantage les conditions retenues, d'autant que les critères proposés dans l'amendement pourraient être contournés

les deux amendements suivants, qui concernent également la défiscalisation des bateaux de croisière. Cet amendement tend à modifier la base éligible, fixée à 20 % des coûts de revient du navire. Cette base éligible étant trop restrictive, il est proposé de la fixer à 50 % afin de permettre au secteur de la croisière de se développer. Quel

C'est une vraie avancée pour les collectivités d'outre-mer ! Mais cet article ne prend pas suffisamment en compte les coûts de construction, qui sont bien plus élevés en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs sur le territoire français, du fait de l'insularité et de l'éloignement. de relever le plafond du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt par logement de 50 000 à 80 000 euros. Quel

de loi de finances étend le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 C du code général des impôts aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines zones des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le présent amendement a pour objet de prévoir la reprise de la réduction d'impôt en cas de non-respect des conditions encadrant l'octroi de l'avantage fiscal au titre de cette nouvelle mesure et de celle, relative aux opérations d'acquisition et réhabilitation de logements de plus de vingt

et qui constituent le prolongement de l'activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif ", telles que " la promotion et l'organisation de congrès, de réunions, la publication d'ouvrages et de revues de nature syndicale, l'exploitation d'un site internet lié à l'activité syndicale, la promotion collective et générale d'un produit

loin. « Les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités. « que les activités pouvant être considérées comme lucratives, ce qui n'apparaît pas illogique. « Les syndicats, dont la gestion est désintéressée et dont l'activité non lucrative est significativement prépondérante, qu'ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicats de la loi de 1884, continueront en outre d'être exonérés d'impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisation foncière des entreprises au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n'excède pas 62 250 euros

tend à aménager le dispositif actuel, qui paraît être source d'insécurité financière pour les entreprises de par sa complexité. De plus, il semble que ce mécanisme crée des effets de seuil préjudiciables. En effet, dans le cas où l'entreprise aurait pour projet de produire dans l'année à venir autant de projets francophones que de projets non francophones, si un seul des projets francophones ne se poursuit pas jusqu'à son terme ou s'il prend du retard et est reporté à l'exercice suivant, alors l'entreprise perd le bénéfice du crédit d'impôt pour l'intégralité des albums non francophones. Certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d'anticiper au moment du dépôt de l'agrément provisoire quels albums précis elles produiront dans l'année à venir. Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l'effet de seuil en indiquant que tout album francophone donne le droit à l'éligibilité d'un album en langue étrangère.

de la part du rapporteur général de l'Assemblée nationale de limiter dans le temps les crédits d'impôt pour les faire correspondre à la loi de programmation des finances publiques, mais il nous semble qu'il a omis un élément essentiel : évidemment, en matière de culture- et je dirai un mot sur le spectacle vivant -, les projets se construisent souvent sur plusieurs années. Il est alors essentiel que les professionnels aient une visibilité pluriannuelle. C'est dans ce sens que le Gouvernement a sous-amendé la proposition du rapporteur général de l'Assemblée nationale en sortant du cadrage général deux crédits d'impôt, dont celui sur les jeux vidéo. C'est là une première source d'étonnement : les studios de développement auraient donc besoin d'une visibilité pluriannuelle- ce que je comprends -, mais pas les producteurs de spectacles Pourtant, les deux dispositifs fiscaux fonctionnent exactement de la même manière, avec notamment une période d'éligibilité commune. La seconde source d'étonnement, c'est que malgré la réussite pleine et entière

Mais il faut rappeler deux éléments : premièrement, alors que l'investissement gouvernemental dans le secteur escomptait 14 millions d'euros en tout, sur la période, on en est à 16,2 millions d'euros, donc bien loin d'une explosion budgétaire deuxièmement, les deux bilans faits par le cabinet Ernst & Young et le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Joël Giraud, sont particulièrement positifs : sur la seule année pleine, le dispositif a concerné 146 très petites, petites ou moyennes entreprises, pour un total de 2 400 dates supplémentaires programmées, 874 projets culturels suivis, soit presque 15 000 représentations, et un chiffre d'affaires représentant presque 40 millions d'euros. Si tous les crédits d'impôt avaient un tel taux d'efficacité, nos finances publiques se porteraient porteraient autrement mieux. C'est pour cette raison qu'il ne nous paraît pas pertinent de revenir sur ce dispositif essentiel, qui a fait ses preuves. Quel

« spectacle vivant ». La durée d'application de ces trois crédits d'impôt jusqu'au 31 décembre 2022 est en cohérence avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, tout en offrant une visibilité suffisante aux professionnels du secteur, point que vous avez vous-même rappelé dans votre intervention.

manque de compétence, j'ai le sentiment que, aussi bien pour créer des jeux vidéo que pour faire du spectacle vivant, il faut laisser du temps au temps. Par ailleurs, les évaluations que j'ai indiquées sont extrêmement pertinentes.

vise à instituer un crédit d'impôt ayant deux objets : d'une part, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; d'autre part, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 euros le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser le e-commerce. Dans les deux cas, il s'agit d'aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique. J'espère que le secrétaire d'État chargé du numérique y sera sensible

Sur ce sujet, vous comprenez que nous partageons la même ambition. Depuis près d'un an et demi, le Gouvernement mène l'initiative France Num à destination des chefs de petite et de moyenne entreprise à travers tout le territoire. Le but est d'apporter des solutions à la fois

Il est plus facile pour une entreprise productrice d'avoir son artiste et sa salle et de mener une petite campagne de promotion, puis de bénéficier du bouche-à-oreille que de déménager et de recommencer son travail de publicité. De fait, il paraît compliqué de conditionner l'accès au crédit d'impôt à un nombre de salles défini.

défavorable sur l'amendement

part de son souhait de procéder à un large passage en revue des crédits d'impôt dédiés à la culture et s'était fixé comme objectif l'évaluation et l'équité entre les secteurs. On ne comprend donc pas bien pourquoi les spectacles d'humour ont été exclus. Le Jamel Comedy Club, qui recèle de nouveaux talents, aimerait bien pouvoir profiter aussi de ce crédit d'impôt.

permettant d'exclure du bénéfice du crédit d'impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d'une jauge supérieure à 6 000 personnes. Le but est de contrer les effets d'aubaine. Enfin, je demande que l'entrée en vigueur de ce crédit d'impôt remanié soit reportée au 1 avril 2019. Maintenir la date du 1 janvier 2019 créerait une insécurité juridique pour les entreprises de spectacles.

qui oeuvrent dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés. L'objet de cet amendement est donc d'étendre le crédit d'impôt spectacle vivant aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.

pénaliserait les entrepreneurs qui parviennent effectivement à faire émerger un artiste- c'est l'objectif même du crédit d'impôt -puisqu'un spectacle ne serait plus éligible s'il venait à être présenté dans des lieux d'une certaine jauge, ce qui

de remplacer le critère négatif d'exclusion des comédies musicales par un critère positif d'inclusion en fonction de la catégorie de spectacle et, enfin, de supprimer la « prime à rester petit

le premier signataire, vise à doubler le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle à hauteur de 60 % de ces dépenses. Est ainsi proposée la création d'un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative à ces produits. Le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition d'une meilleure maîtrise de leur utilisation. Le développement de solutions alternatives est également un enjeu majeur pour l'agriculture française, qui doit répondre au défi alimentaire, tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse, par ailleurs, les collectivités, ainsi que les particuliers, qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires

Les produits de biocontrôle bénéficient déjà de soutiens et de régimes dérogatoires par rapport au droit commun. Je pense notamment aux procédures accélérées d'évaluation et d'instruction des demandes,

en la matière ! La situation est relativement dramatique. Les mauvaises herbes se multiplient dans les cultures et l'on ne maîtrise plus rien à force de retirer des matières actives en l'absence de moyens de substitution. J'entendais hier un bruit infernal dans le jardin du Luxembourg, où l'on désherbait au chalumeau,

qui reprend avec quelques modifications une préconisation du rapport de juin 2018 de M. Martial Bourquin, fait au nom de la mission d'information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays. Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit d'impôt recherche à un engagement de maintien de l'activité de l'entreprise sur le territoire national pendant un délai de cinq ans à compter du 1 janvier de l'année suivant celle où l'entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. En effet, pour reprendre un constat que nous avons fait il y a plusieurs années et qui est d'une actualité saisissante, le Gouvernement explique tous les jours que les caisses de l'État sont vides et qu'il est indispensable de faire des économies, mais commençons par voir si l'argent dépensé l'est utilement, et regardons là où l'on n'a pas l'habitude de regarder ! De ce point de vue, le crédit d'impôt recherche est tout à fait exemplaire. Il pèse un poids considérable : son montant, 6 milliards d'euros, en fait l'une des principales niches fiscales depuis plusieurs années.

mais aussi nationaux, qui bénéficient du CIR sans exercer leur activité sur le territoire national. Ce crédit d'impôt doit s'accompagner d'une contrepartie, avec une présence suffisante en France pour permettre un juste retour pour la collectivité de l'effort fiscal consenti. L'amendement n° II-828 rectifié,

un engagement de maintien de l'activité de l'entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1 janvier de l'année suivant celle où l'entreprise a exposé ses dépenses de recherche. À défaut d'assurer le respect de cette condition de durée, le dispositif organise un mécanisme de reprise de l'avantage fiscal octroyé. Cette mesure était l'une des recommandations

Ainsi, le dispositif en lui-même ne génère pas d'effet d'aubaine ou d'optimisation fiscale. D'un point de vue plus technique et juridique, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait considérer que le fait de conditionner le bénéfice du crédit d'impôt à un engagement de maintien de l'activité de l'entreprise sur le territoire national pendant un certain délai est contraire à la liberté d'établissement. Je vous renvoie ainsi à l'arrêt Fournier du 10 mars 2005, dans lequel répondant à une question préjudicielle, a estimé que réserver le bénéfice du CIR à des opérations de recherche uniquement réalisées en France était contraire au droit communautaire. Enfin, plus particulièrement sur l'amendement n° II-828 rectifié, je me permets de rappeler que le crédit d'impôt recherche est un dispositif

Monsieur Savoldelli,

la commission des affaires économiques a souligné l'importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l'enjeu stratégique aujourd'hui considérables de la normalisation.

au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, le CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel en 2012 dans son rapport au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l'économie, alors Actuellement, aux termes de l'article 244 B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Cet amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

En effet, à l'intérieur des dépenses de normalisation sont pris en considération les éléments de salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation, les autres dépenses liées à cette participation, prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires, ainsi que les dépenses effectuées, notamment par les chefs d'entreprise, pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à raison d'un forfait de 450 euros par jour. Par ailleurs, je rappelle qu'il existe des aides financières non fiscales destinées à couvrir les frais liés à la participation aux réunions des organes européens de normalisation par les organisations professionnelles représentant les entreprises. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'élargir l'assiette des dépenses de normalisation ou d'augmenter leur montant,

compte tenu du poids économique et de l'enjeu stratégique aujourd'hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation à l'échelon tant national qu'européen ou international. Dans ce contexte, la commission a regretté que le régime actuel, défini à l'article 244 B du code général des impôts, limite le bénéfice du CIR aux seules dépenses concernant les salariés et dirigeants de l'entreprise, ne prenne pas en considération les frais liés à la rémunération de consultants extérieurs engagés par l'entreprise. Cette solution est défavorable aux PME, qui n'ont souvent pas les moyens humains de faire participer leur propre personnel salarié aux travaux de normalisation, et peuvent ressentir le besoin de recourir à une expertise extérieure. Cet amendement vise donc à élargir également aux dépenses engagées pour la rémunération et la participation des personnes autres que les salariés de l'entreprise le bénéfice du CIR lorsque celles-ci représentent cette société dans les instances de normalisation, à concurrence d'un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de présence dans ces instances.

Je rappelle que la méthode de calcul de la valeur locative a été créée à l'origine pour favoriser les établissements industriels. Ils ne sont pas redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et bénéficient d'un abattement au titre de la cotisation foncière des entreprises, toute requalification d'un établissement industriel en local professionnel n'est pas favorable à l'entreprise, d'autant que les valeurs locatives des locaux professionnels ont été révisées.

notamment, les établissements des entreprises de bâtiment qui réalisent des ouvrages en atelier et qui vont les poser sur des chantiers, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage. L'article 56 du projet de loi de finances pour 2019 donne une nouvelle définition des établissements dits « industriels » au regard de l'article 1500 du code général des impôts, le CGI. Cette disposition tente de légaliser l'absence d'une telle définition dans le CGI et, ainsi, de mettre fin au flou entourant entourant les impositions locales de nombreux établissements. Faute de définition légale de la notion d'établissement industriel, l'administration en avait fait une interprétation extensive, s'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement

portant sur trois ans, la trésorerie des entreprises est fortement handicapée. D'autre part, dans un contexte économique qui reste difficile, les entreprises du bâtiment, qui ont jusqu'à présent privilégié l'emploi, se posent aujourd'hui la question de savoir si la fabrication en France mérite d'être poursuivie. Enfin, on ne peut qu'être surpris du décalage existant entre certains voisins européens, qui exportent leurs menuiseries avec le soutien de l'État et des fonds européens, et la France qui, tout en améliorant la compétitivité de ses entreprises, laisse ces dernières subir les conséquences dommageables d'une fiscalité complexe et confiscatoire.

Lavarde. Je croyais que les dispositions du texte initial étaient le résultat de négociations menées en amont entre le Gouvernement et un certain nombre d'associations. Toutefois, certaines associations, qui n'étaient peut-être pas présentes autour de la table, sont venues m'expliquer qu'elles contestaient ce point d'équilibre.

L'objet de cet amendement, à défaut d'exclure purement et simplement les activités du bâtiment de la notion d'établissement industriel, est de préciser le montant minimal des matériels, outillages et installations techniques. En effet, les activités potentiellement visées par la notion d'établissement industriel sont importantes et variées. Selon l'activité, le recours aux moyens techniques est plus ou moins important. Or fixer un montant unique ne tenant pas compte du caractère capitalistique de chacune des activités ne résout pas la difficulté et crée une inégalité entre les contribuables. Ainsi, il est proposé de renvoyer ce montant minimal de moyens techniques à un décret qui fixerait ce chiffre activité par activité.

à la question du bon niveau d'information et de la juste définition des seuils. Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de supprimer la légalisation de la définition des établissements industriels, ainsi que le seuil de matériels et outillages en dessous duquel un local ne serait plus qualifié d'établissement industriel. Vous proposez également de remplacer la remise d'un rapport relatif au changement de méthode d'évaluation de ces établissements par celle d'un nouveau rapport portant sur les conséquences de la mise en oeuvre d'un seuil de matériels et outillages de 300 000 euros ou de 500 000 euros, en deçà duquel les terrains et bâtiments ne seraient pas qualifiés d'établissements industriels. Nous ne sommes pas favorables à cet amendement. Il n'existe pas aujourd'hui de définition des établissements industriels au sens foncier dans le code général des impôts. La légalisation à droit constant de cette construction purement jurisprudentielle a pour objet d'en stabiliser la définition et d'empêcher toute nouvelle interprétation extensive par le juge. Cette mesure aura donc pour effet de sécuriser les impositions à venir des acteurs économiques- un objectif important pour vous, monsieur le rapporteur général -et d'éviter de nouvelles requalifications issues d'interprétations erronées de la notion d'établissement industriel.

Concernant le seuil, il avait été initialement fixé à 300 000 euros par le Gouvernement. L'Assemblée nationale, après consultation, l'a porté à 500 000 euros. euros. Le Gouvernement continue de considérer qu'il s'agit d'un seuil raisonnable pour caractériser l'importance des moyens techniques servant à qualifier un local d'établissement industriel. Il permet notamment de sécuriser la qualification des locaux utilisés par les PME, tout en limitant les impacts pour les collectivités. Nous reconnaissons qu'il n'est pas possible actuellement pour l'administration de simuler les conséquences de la mise en oeuvre de ce seuil. C'est pourquoi la détermination d'un seuil proche de la jurisprudence actuelle permet d'éviter d'exclure un nombre trop significatif de locaux de la catégorie des établissements industriels, et assure une certaine sécurisation, dans la continuité de la jurisprudence. Vous souhaitez enfin remplacer la campagne déclarative prévue à l'article 56 par une campagne déclarative limitée aux seuls propriétaires des bâtiments et terrains affectés à une activité entrant dans le champ

que l'administration pourra déterminer les effets d'un changement potentiel de méthode d'évaluation des établissements industriels. C'est pourquoi un amendement en ce sens avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement. Cette démarche permettra de déterminer les effets d'un potentiel changement des modalités d'évaluation des établissements industriels. Ce n'est qu'une fois ce travail réalisé, et avec un rapport remis sur ce sujet par l'administration au plus tard le 1 avril 2020, que les décideurs publics pourront, en toute connaissance de cause, engager une concertation pour décider, le cas échéant, de faire évoluer la méthode d'évaluation des locaux industriels. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° II-745, monsieur le rapporteur

amendement vise à renforcer le lissage dans le temps des conséquences d'une requalification en établissement industriel.

aux forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'aux renseignements territoriaux qui, depuis deux jours, agissent avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid, en particulier devant les lycées de nos territoires. Des photos prises au commissariat de Mantes-la-Jolie créent la polémique. Cette polémique est indigne, alors que les raisons et les conditions d'interpellation des jeunes concernés ne sont jamais mises en avant. Lorsque les interpellations ont été réalisées, des violences extrêmement importantes étaient en

celle dans laquelle nous sommes habitués à faire des cérémonies patriotiques. Dans des délais très courts, les jeunes ont été redirigés vers d'autres commissariats, et j'insiste sur le fait que des émeutes ont été évitées, qu'il n'y a eu aucun blessé, aucune plainte, aucune faute et que tout s'est réalisé sous le contrôle permanent du juge qui était présent. Dans ces conditions, je réitère- je souhaite que la Haute Assemblée puisse le faire avec moi -mon total soutien aux forces de l'ordre,